Je vous rappelle que, dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes ; l’auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répartie, pour une minute.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’année 2024, qui n’est pas encore terminée, a été marquée par des records de pluviométrie. Cette situation est exceptionnelle et même atypique, puisqu’elle intervient après plusieurs années de sécheresse dans une large partie du territoire hexagonal. Gouverner, c’est prévoir et c’est donc anticiper. Nous avons la chance au Sénat de disposer d’une délégation à la prospective dont c’est précisément la mission. Son rapport d’information intitulé, remis à la fin de l’année 2022 et dont j’étais corapporteur, a posé un diagnostic clair et implacable, confirmé par la mission conduite l’année dernière par nos collègues Rémy Pointereau et Hervé Gillé les cycles hydriques se modifient sous l’effet du changement climatique, faisant alterner des épisodes de fortes précipitations au printemps et à l’automne, et des épisodes prolongés chauds et secs en été, parfois aggravés par des sécheresses hivernales. Tordons le cou à une idée fausse : nous n’aurons pas globalement moins d’eau. En effet, l’eau est une ressource renouvelable et le réchauffement climatique conduit à s’exposer à plus de précipitations puisque la quantité d’eau qui s’évapore des océans a tendance à retomber en plus grande quantité sur les terres émergées.

Nous attendons les résultats de l’étude Explore2 qui devraient affiner ces prévisions et en préciser la géographie. Mais une chose est sûre : tous les territoires, même au nord du pays, seront touchés. Le récent épisode espagnol en est un exemple concret. Dans Dans ce contexte, ne rien faire serait catastrophique. Gérer l’eau, et la domestiquer, est consubstantiel à la civilisation. Il convient non seulement de se prémunir contre les inondations, mais aussi de sécuriser notre approvisionnement en eau potable, de savoir l’utiliser pour l’industrie, pour la production d’énergie ou encore pour l’agriculture. Au passage, notons que l’agriculture irriguée ne représente que 10 % des surfaces agricoles, soit moins de 3 millions d’hectares. Bien entendu, il faut tirer les leçons du passé et ne pas se lancer dans des aménagements hydrauliques néfastes à l’environnement et à la biodiversité. Nous disposons désormais des connaissances nécessaires et d’un cadre juridique très exigeant pour ne pas tomber dans les travers de tels aménagements.

Sachons appliquer avec discernement le principe de précaution, en n’opposant pas l’environnement à l’activité économique et en essayant de faire dialoguer les différentes parties prenantes.

commissions locales de l’eau. Les sécheresses successives rendent ce modèle du consensus de plus en plus fragile, mais il n’y a pas d’autre voie que celle du dialogue et de la concertation, sous réserve bien évidemment que les différents acteurs s’engagent de bonne foi. 2024 nous offre un répit, qui ne doit pas nous faire oublier que les restrictions d’eau pourront revenir très vite. Elles n’ont d’ailleurs pas disparu, cette année, sur la totalité du territoire.

réaliser de nouvelles retenues de l’eau venant des Pyrénées, là où c’est possible, en plus des barrages de Vinça ou de l’Agly. Nous devrons développer les retenues collinaires dans les exploitations agricoles, en réduisant la durée des procédures d’autorisation et en les simplifiant, ce qui diminuera aussi les coûts. le coût des études préalables est bien souvent plus élevé que celui des travaux ! Il conviendra aussi de pratiquer davantage la réutilisation des eaux usées traitées, notamment dans la zone littorale, pour des usages autres que l’approvisionnement en eau potable.

Pour conclure, madame la ministre, mes chers collègues, il n’est pas tenable de faire reposer l’essentiel de la stratégie pour l’eau des Pyrénées Orientales sur des efforts d’économie. Beaucoup a déjà été fait en la matière. Les communes littorales gèlent le développement touristique pour ne pas davantage solliciter la ressource en période d’étiage.

Ne soyons pas lents ou timides. Des solutions existent. Arrêtons de multiplier les études et les comités Théodule. N’attendons plus pour agir, car il y a urgence. Les pluies de 2024 ne nous ont donné qu’un court répit. La parole

Jaubert. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, malgré une pluviométrie abondante au printemps et au début de l’été dernier, vingt et un départements ont tout de même dû faire face à des restrictions importantes imposées par les préfectures. Ces mesures montrent bien qu’une gestion durable de l’eau ne peut plus dépendre uniquement des conditions saisonnières, mais qu’elle nécessite des réponses structurelles. Nous le savons tous, la gestion de l’eau est une question cruciale et l’été 2024 n’a fait que renforcer cette réalité, notamment en Gironde, département qui a été placé en état de crise en raison de la baisse du débit des cours d’eau. Les périodes de restriction sont devenues la norme et non plus l’exception. Durant l’été dernier, les limitations d’usage ont affecté l’arrosage des jardins, l’irrigation des cultures et même certaines activités économiques. Or ces mesures ne sont que des solutions temporaires qui ne constituent ni une réponse d’envergure ni une réponse de long terme. La gestion de l’eau peut notamment être appréciée au regard de la vétusté de nos infrastructures et de l’inefficacité de notre système de distribution, où chaque goutte compte désormais. Je souhaite ici poser une question essentielle : comment peut on accepter que plus de 20 % de notre eau potable se perde chaque jour en raison de fuites ? Ce chiffre, bien trop élevé, n’est pas seulement une donnée technique. Il est aussi le reflet d’années de sous investissements dans nos réseaux d’eau. La modernisation de nos canalisations,

Dans la continuité de ce qui avait été proposé par Nathalie Delattre et le groupe du RDSE lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, je suggère la création d’un fonds bleu de solidarité pour soutenir la rénovation des réseaux d’eau en France.

Si ce transfert budgétaire est maintenu dans les années à venir, d’autres sources de financement devront être envisagées, comme l’établissement de contributions fondées sur la consommation d’eau, sur le modèle de l’ancien fonds national pour le développement des adductions d’eau. Ce fonds, financé en partie par une taxe sur les paris du PMU et par une redevance sur l’eau potable, pourrait servir de référence. Une fois financé, ce fonds bleu pourrait être redistribué prioritairement aux communes et aux syndicats dont les infrastructures sont les plus dégradées. En Gironde, par exemple, de nombreux syndicats de petite taille peinent à assurer l’entretien de leur réseau, en comparaison de ce qui se fait dans les grandes villes comme Bordeaux. En partenariat avec les agences de l’eau, les conseils départementaux doivent également apporter un soutien technique aux plus petites communes pour cibler les rénovations

Il faudra aussi sensibiliser toujours plus la population sur les usages non essentiels de l’eau potable, que l’on doit réserver à la consommation humaine et à la préservation de la santé publique.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les événements dramatiques survenus récemment en Espagne illustrent de façon tragique les conséquences dévastatrices du dérèglement climatique sur le cycle de l’eau. Les sécheresses et les inondations extrêmes qui se succèdent à travers l’Europe révèlent l’ampleur de la crise hydrique qui nous menace.

qui prennent la forme d’un assèchement des sols, d’une baisse drastique du niveau des nappes phréatiques et de tensions exacerbées entre les différents usages. L’intensité des périodes de sécheresse que nous avons connues ces dernières années et leur fréquence accrue percutent sérieusement notre gestion de cette ressource vitale. mettre en œuvre une politique de régulation et de partage de l’eau à la hauteur des enjeux. L’heure est venue de repenser en profondeur notre modèle de gestion de l’eau. C’est pourquoi j’attire votre attention, ce soir, sur trois sujets qui méritent réflexion : les mécanismes de concertation pour la gestion de l’eau,

Cette construction, autorisée par la préfecture, a été réalisée sans étude préalable sérieuse et sans aucune consultation des parties concernées. Il s’agit d’une question environnementale, mais également d’ordre public : comment préviendrons nous la montée des tensions liées à l’eau alors que celle ci se raréfie ?

Une première solution pour réduire la fréquence des conflits d’usage serait de ne pas gaspiller la ressource. Pourtant, certaines de nos communes voient jusqu’à 30 % de leur eau potable se perdre au travers de fuites dans les réseaux de distribution.

Dans le contexte actuel de sécheresses répétées, où nous demandons des efforts considérables à la population pour réduire sa consommation, ce niveau de rendement est loin d’être suffisant. Les collectivités locales sont en première ligne face au défi de l’approvisionnement. Toutefois, elles peinent à faire face à la complexité technique et aux coûts élevés des travaux nécessaires pour moderniser leurs infrastructures de distribution et d’assainissement. Le Gouvernement a bien pris connaissance de cette problématique, qui est identifiée dans le plan Eau. Au total, 170 points noirs ont été répertoriés par les services de l’État, soit 170 communes, intercommunalités ou syndicats où 50 % de la ressource est perdue dans les canalisations : un litre sur deux est

ailleurs, l’eau est particulièrement bon marché en France par rapport à d’autres pays européens. Ce faible coût, tout en étant un facteur de justice sociale, envoie également un signal ambivalent quant à la valeur de la ressource, dont la rareté se fait de plus en plus sentir. Actuellement, dans notre pays, le prix moyen de l’eau potable est d’environ 3,56 euros par mètre cube, soit 11 % de moins que la moyenne européenne. Ce tarif ne reflète pas l’ensemble des efforts nécessaires pour garantir à chacun un approvisionnement en eau propre et potable. Ces efforts, déjà coûteux

Alors que vous promouvez, madame la ministre, la sobriété comme une valeur cardinale, la question du prix de la ressource sera t elle à l’agenda ? Autrement dit, si tant est que « l’eau paie l’eau », le coût des travaux nécessaires pour moderniser notre système d’approvisionnement sera t il répercuté sur les tarifs ? Madame la ministre, lors de votre dernière audition par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, que j’ai l’honneur de présider, vous avez évoqué le besoin de repenser la gestion de la ressource. Aujourd’hui, en portant à votre attention ces pistes de réflexion, je vous propose d’aller plus loin,

Ces variations, aléatoires, d’une année sur l’autre confortent l’idée que nous devons renforcer les moyens de l’État et de ses établissements publics pour élaborer des méthodologies fiables de prévision des disponibilités

avoir du sens. Nous devrons renforcer les moyens de nos services publics pour fonctionner à cette échelle et pour améliorer ainsi la prévention des risques. Les défis sont devant nous.

Au lieu de cela, le Gouvernement les maintient au niveau de 2024 dans le projet de loi de finances à venir. Si nous nous réjouissons que les communes qui le souhaitent

je veux préciser que, si nous améliorons nos connaissances sur l’eau, sa gestion et son partage, celle ci peut aussi devenir une opportunité économique, notamment énergétique. Nous pouvons profiter de cet élément naturel pour soutenir les énergies renouvelables, avec la production hydroélectrique et les stations de transfert d’énergie par pompage (Step) et aboutir ainsi à une stratégie nationale ambitieuse, territorialisée, nous

Cette situation nous impose de repenser en profondeur notre rapport à l’eau et d’adopter une approche globale et cohérente. Premièrement, nous devons faciliter la pénétration naturelle de l’eau dans nos sols. C’est la clé de voûte d’une gestion durable de notre ressource, les nappes phréatiques sont nos réserves naturelles et leur recharge doit être notre priorité. Concrètement, cela signifie repenser nos pratiques d’aménagement du territoire. En Gironde, certaines collectivités ont déjà mis en place des projets pilotes prometteurs.

de territoire. Ils doivent être non pas une solution de facilité, mais un outil parmi d’autres dans une stratégie globale. Quand ils sont bien conçus et bien intégrés, ces ouvrages multi usages permettent de stocker l’eau en période d’abondance pour la restituer lors des périodes de stress hydrique.

doit être développée quels que soient les usages pour engager l’ensemble des parties prenantes sur des objectifs communs. Troisièmement, nous devons impérativement développer une stratégie de sobriété hydrique. Cela passe par plusieurs leviers : une meilleure gestion des eaux pluviales, notamment en milieu urbain,

est donc essentielle pour assurer le ressuyage des sols, leur régénération naturelle et l’évacuation contrôlée des eaux pluviales. Cela permettrait de mieux gérer l’eau à l’échelle du territoire, de limiter l’imperméabilisation des sols et de garantir une évacuation contrôlée des eaux pluviales, notamment en période de fortes pluies. Une telle approche doit être systématiquement intégrée dans les documents d’urbanisme afin de structurer une gestion durable et préventive à l’échelle de chaque commune. Nous l’avons vu également dans le Pas de Calais : la qualité des réseaux hydrologiques est essentielle et doit nous intéresser prioritairement. Mes chers collègues, la gestion de l’eau est une question non plus technique, mais politique, au sens général : c’est un défi de société qui nécessite une approche systémique. Les événements de l’été 2024 nous ont montré que nous devions agir vite, mais surtout intelligemment, et mobiliser tous les moyens nécessaires, notamment en matière de prévention.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, face au caractère désormais irréversible des mutations entraînées par le changement climatique, nous sommes contraints d’accélérer nos transitions et d’adopter une stratégie d’atténuation et d’adaptation. Les défis liés aux sécheresses répétées et aux tensions croissantes entre les différents usages de l’eau

de précipitations, suivis, par endroits, d’épisodes pluvio orageux. À l’inverse, certaines zones, comme le Bassin parisien, la Champagne Ardenne, les Hauts de France ou le Massif central, ont connu des pluies diluviennes et des orages violents, ces événements provoquant inondations et importants dégâts – nous en savons quelque chose,

vivre… Délocalisation des bassins de production, déplacements de populations, concurrence pour le foncier et pour l’accès à la ressource en eau : ces phénomènes créent des tensions et des arbitrages doivent être faits. La gestion de l’eau constitue un sujet crucial, à l’échelle des territoires. actionnés et différents aménagements sont possibles pour assurer une gestion plus efficiente de cette ressource, et notamment des excédents d’eau : zones tampons,

permet de stocker l’eau de surface quand celle ci ruisselle – je vous épargne le raisonnement, vous le connaissez par cœur : Mme la ministre nous a même expliqué qu’elle avait eu l’occasion,

Hélas ! les tensions autour des réserves d’eau se sont accentuées ces dernières années, entre besoins agricoles et préoccupations écologiques notamment – ne faisons pas l’erreur d’opposer les deux À cela s’ajoutent des obstacles économiques et des exigences environnementales, ainsi que la complexité et la lenteur des démarches administratives – en particulier pour nos agriculteurs. L’eau est un bien commun dont l’usage doit être équilibré ; mais il est indispensable de nous adapter vite et d’éviter les oppositions de principe. Les retenues collinaires sont des solutions efficaces et durables de gestion de l’eau.

Pour relever ce défi, cinq conditions me paraissent essentielles. Premièrement, il faut évaluer. Il est impératif de disposer d’une connaissance la plus fine possible de la ressource en eau souterraine et superficielle sur tous nos territoires de plaine, de demi montagne et de haute montagne. Tous les moyens de prospection et de recherche doivent être mis en œuvre à cet effet. Deuxièmement, il faut protéger. Après avoir évalué la quantité disponible, il est essentiel d’assurer la qualité de l’eau selon les usages envisagés : les normes requises sont différentes selon que l’eau est destinée à la consommation humaine, à l’assainissement, à l’irrigation, au stockage, aux loisirs, au thermalisme, etc. Dans une optique d’anticipation des périodes de sécheresse futures, des mesures s’imposent visant la sobriété pour tous les usages.

de solliciter économies et rationalisation quand le rendement est si déficitaire. Aussi des efforts doivent ils porter sur le diagnostic des réseaux et sur la programmation des travaux nécessaires pour colmater les fuites et optimiser le rendement.

permet de sécuriser la ressource en eau potable et de compléter les actions de sobriété et d’efficience des collectivités. Mais cette solidarité peut et doit s’exprimer

n’est pas tabou… –, permettent de stocker l’eau de pluie, peuvent prévenir les inondations et limitent l’érosion des sols. Après avoir évalué, protégé, rationalisé, connecté et stocké, nous devons tous agir en responsabilité et en solidarité

d’améliorer à la fois la sobriété de nos usages et notre résilience face à l’évolution de la ressource.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce débat inscrit à notre ordre du jour par le groupe Les Républicains nous conduit à nous interroger sur la gestion de l’eau : comment préserver cette ressource ? Je me félicite que nous puissions débattre de ce sujet. Cette thématique nous oblige, en tant que citoyens, mais surtout en tant que législateur. Il n’est pas vain de rappeler combien la gestion de l’eau est vitale, non seulement pour l’avenir de notre planète, mais aussi pour celui de l’espèce humaine. effet une ressource indispensable pour notre santé, pour nos écosystèmes, pour notre agriculture et pour notre économie, mais, trop souvent, nous prenons cette ressource pour acquise. En plus, nous la croyons éternelle… Débattant de ce sujet, nous ne saurions faire l’économie de la question du changement climatique. L’accès à l’eau et la gestion de cette ressource demeurent des enjeux majeurs dans le contexte du réchauffement climatique.

ainsi que les dommages sociétaux qui en découlent ». C’est ainsi que les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations et les sécheresses, sont de plus en plus fréquents et intenses. J’en veux pour preuve la fermeture actuelle de plusieurs écoles en Guyane en raison de la sécheresse et d’un niveau exceptionnellement bas du fleuve Maroni, les embarcations qui transportent les élèves ne peuvent plus circuler. Les habitants du Maroni sont ravitaillés grâce à un pont aérien mis Cet été encore, près de quarante départements ont été concernés par des mesures de restriction d’eau, la sécheresse ayant épuisé les ressources en eau plus tôt que d’habitude. Dans le sud est de la France comme en Bretagne, région habituellement épargnée, on a ainsi observé une baisse significative du niveau des nappes phréatiques. Nous devons être lucides : les besoins en eau dépassent très régulièrement notre capacité d’approvisionnement et ce phénomène n’est pas près de s’inverser. Selon de nombreuses études, il apparaît qu’à l’horizon de 2050 les débits annuels moyens pourraient diminuer de 10 % à 40 % ; la vitesse de recharge des nappes de 10 % à 25 %,

En effet, selon la Commission européenne, plus de 40 milliards de mètres cubes d’eaux usées sont traités chaque année dans l’Union européenne, dont moins de 1 milliard seulement En France, 99 % des eaux usées sont rejetées dans le milieu naturel après leur passage en station d’épuration. Le plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau a ainsi prévu la réalisation de 10 % d’économies d’eau d’ici à 2030.

pour atteindre cet objectif ? Je veux également évoquer la nécessité d’améliorer la gestion des réseaux d’eau. L’ancienne présidente de communauté d’agglomération que je suis connaît les conséquences des fuites d’eau, provoquées par le vieillissement de nos infrastructures. Chaque année, près de 1 milliard de mètres cubes d’eau sont perdus, soit l’équivalent de 20 % de la production nationale d’eau potable. Autrement dit, pour cinq litres d’eau mis en distribution, un litre retourne directement au milieu naturel sans passer par le consommateur. Aussi, en tant qu’Ultramarine, ne puis je aborder cette question des réseaux de distribution sans avoir une pensée pour mes compatriotes guadeloupéens. Depuis des mois, une partie des habitants de leur île est privée d’accès à l’eau du robinet à cause de l’état désastreux des réseaux. À maintes reprises, mes collègues guadeloupéens ont interpellé le Gouvernement sur cette question. Je vous demande, madame la ministre, de soutenir financièrement l’ensemble des collectivités et des syndicats mixtes, particulièrement en zone rurale, dans la perspective d’une amélioration des réseaux de distribution. Quels engagements pouvez vous prendre en la matière ? Il ne fait aucun doute que les initiatives bien qu’elles démontrent notre volonté d’innover, ne parviendront pas à elles seules à stopper l’hémorragie. Mes chers collègues, j’estime que désormais chaque goutte compte. Il est crucial de renforcer les campagnes de sensibilisation menées auprès du grand public, et surtout à destination de la jeune génération. La rareté de l’eau nous impose de changer de paradigme ; chacun, où qu’il se trouve, doit jouer un rôle dans la préservation de cette ressource vitale. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, beaucoup l’ont dit avant moi, les tensions politiques et sociales s’exacerbent sur le sujet de l’eau depuis maintenant de nombreuses années, car cette ressource va devenir de plus en plus rare.

Nous avons perdu 32 milliards de mètres cubes d’eau ; nous pourrions en perdre 50 milliards supplémentaires dans les années qui viennent, sous l’effet du réchauffement climatique. Se pose également la question centrale – j’y reviendrai – de la qualité

vertes, il suscite lui aussi beaucoup d’interrogations. La région Bretagne a réaffirmé sa volonté d’être aux côtés de l’État pour le copiloter et pour cofinancer les projets de territoire des huit baies concernées. En 2025, nous serons à mi parcours du plan

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le sujet qui nous réunit ce soir, la gestion de l’eau, occupera très certainement une part croissante de nos travaux dans les années à venir. La raison en est aussi simple qu’implacable

à préparer sans tarder notre résilience hydrique. Deux constats issus de cette étude suffisent à qualifier l’urgence : premièrement, la ressource en eau renouvelable a diminué de 14 % au cours des quinze dernières années

anticipation, pour éviter que les sécheresses à répétition et les stress hydriques plus intenses ne prennent au dépourvu les territoires les plus fragiles ; concertation, pour prévenir les conflits d’usage qui mettent à mal le vivre ensemble, afin d’élaborer de manière collective un nouveau « contrat social de l’eau

d’agences de l’eau, puissants organes de mutualisation financière, de solidarité horizontale et d’investissement dans les réseaux et dans la résilience hydrique ; enfin, d’une démocratie de l’eau, qui vit au sein de multiples structures, sans doute trop nombreuses, depuis le comité de bassin jusqu’aux commissions locales de l’eau. La structure est robuste. Malgré des critiques justifiées, elle a permis à notre pays de traverser plusieurs crises. Il nous faudra néanmoins la consolider face à l’intensité croissante des phénomènes climatiques extrêmes et la rendre plus efficiente encore.

rigueur oblige, mais il devrait reprendre à compter de 2026 pour atteindre les 475 millions d’euros annoncés en 2023. À ce titre, on ne peut que déplorer, madame la ministre, le prélèvement sur les recettes des agences de l’eau à hauteur de 130 millions d’euros

Nous devons être meilleurs dans la réutilisation des eaux usées traitées et dans la sécurisation de l’eau nécessaire à notre souveraineté agricole. La sobriété des usages doit être élevée au rang de priorité et les acteurs doivent être accompagnés dans leur recherche de performance hydrique accrue. La facture d’eau doit aussi mieux refléter la rareté de la ressource au travers d’un signal prix repensé et réaffirmé. Le principe pollueur payeur doit mieux imprégner notre gestion de l’eau, car il devient de plus en plus complexe et onéreux de traiter les micropolluants nouveaux qui affectent la qualité de la ressource et mettent en danger la biodiversité aquatique. La conciliation des différents usages de l’eau aux périodes critiques doit être renforcée au travers d’instances de concertation, de modalités de partage équitable entre tous les acteurs et d’un juge de paix en cas de blocage persistant. À la lumière de ces éléments, mes questions sont donc simples, madame la ministre : quels seront le format et les objectifs de la grande conférence nationale sur l’eau annoncée par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale ? Quand sera t elle lancée ? Qui y participera et quels seront les débouchés législatifs

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, si cet été a été particulièrement pluvieux, les signes de tension hydrique se sont multipliés mettant en lumière l’urgence d’une gestion de l’eau adaptée aux défis de demain. Notre climat tempéré, historiquement généreux en pluies, semble aujourd’hui ne plus suffire à garantir une ressource en eau abondante et accessible pour tous.

l’avenir. Celles ci doivent permettre à la France de faire face aux enjeux grandissants liés à la gestion de cette ressource précieuse. Le changement climatique bouleverse notre cycle de l’eau les précipitations irrégulières, les sécheresses prolongées ou encore les crues soudaines sont autant d’événements qui deviennent la norme et fragilisent l’équilibre naturel de nos réserves. Ce constat est bien entendu préoccupant, mais des solutions existent : avec des efforts notables, une gestion plus durable de la ressource est possible.

Envisager des retenues d’eau multi usages pour capter les précipitations hivernales pourrait aider, par exemple, à pallier le manque d’eau en été. Investir dans des solutions naturelles comme la restauration des zones humides, des prairies et des forêts renforcerait la recharge des nappes phréatiques et limiterait le ruissellement.

En effet, ce secteur essentiel pour notre économie et notre souveraineté alimentaire absorbe près des deux tiers de notre ressource en eau, ce qui en fait un acteur clé dans la gestion durable de cette ressource. Bien que des techniques avancées comme le goutte à goutte soient encouragées pour améliorer l’efficacité de l’irrigation, il est nécessaire – j’insiste sur ce point – de repenser les systèmes de culture pour réduire durablement la consommation d’eau. Évidemment, les changements impliquent des efforts financiers. L’augmentation des budgets des agences de l’eau permettrait de renforcer la résilience collective de nos territoires et de soutenir davantage les projets d’infrastructure et de préservation de l’eau. Enfin, mes chers collègues, n’oublions pas le rôle fondamental de l’éducation. En tant qu’ancien professeur, je mesure l’importance de l’apprentissage pour préparer notre société de demain. La sensibilisation des publics de tous âges à la valeur de l’eau et à sa préservation est essentielle. En mobilisant chaque citoyen, nous pourrons construire un modèle de gestion de l’eau capable de répondre aux défis futurs. Notre responsabilité est d’assurer à nos territoires un accès durable à l’eau, aujourd’hui et pour les décennies à venir, afin que les générations actuelles et futures ne connaissent pas la pénurie. Le tableau est complexe, mais non apocalyptique. La France peut gérer son eau avec intelligence et anticipation, à condition de mettre en œuvre les transformations nécessaires et de prendre des décisions courageuses. Les recommandations de notre rapport sénatorial offrent une feuille de route ambitieuse, mais réaliste, pour atteindre cet objectif. Ensemble, œuvrons pour un avenir où l’eau restera une ressource accessible à tous.

l’objectif est d’améliorer nos connaissances sur ces pollutions et d’agir pour les réduire. À cet égard, trois éléments sont attendus dans le droit fil du plan Eau et de la stratégie Écophyto : un arrêté de définition des points de captage sensibles, un guide à destination des préfets comportant des règles de gestion en fonction des différents cas de figure, et des outils financiers d’accompagnement de changement des pratiques. Le deuxième chantier est la mise en œuvre du plan d’action pour l’eau et l’assainissement dans les territoires ultramarins, que nous avons évoqué avec Mme Phinera Horth.

C’est pourquoi, en parallèle des mesures du plan Eau visant à stabiliser les volumes consacrés à l’irrigation, des réserves de substitution pourront être construites dans les territoires qui sont structurellement en déséquilibre.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis que le groupe Les Républicains ait été à l’origine de ce débat sur la gestion de l’eau, un sujet majeur pour notre avenir. La richesse de nos échanges témoigne de l’importance de cette thématique.

les Pyrénées Orientales, mon cher Jean Sol – et les nappes phréatiques sont à leur plus haut niveau. Cet état des ressources n’est peut être qu’un répit, mais cette situation favorable doit nous permettre de relativiser les prédictions de catastrophes planétaires liées à la pénurie d’eau. Il faut donc anticiper et faire preuve de pragmatisme pour nous adapter au changement climatique : retenir l’eau quand elle est abondante afin de l’utiliser l’été, l’été, créer des bassins d’orage, rehausser les barrages existants pour écrêter les crues et faire face aux inondations. Mon collègue Hervé Gillé et moi même avons récemment présenté un rapport sur la gestion durable de l’eau

elles ont permis de lutter contre la pollution et de concilier les besoins en eau des collectivités locales, de l’agriculture et de l’industrie. Malheureusement, la politique de l’eau est devenue illisible et complexe.

qu’elle mobilise bien trop d’acteurs. Aux côtés des acteurs présents parce qu’élus, on trouve en effet pléthore d’acteurs nommés, d’experts ou d’associations, qui n’aident pas toujours à la compréhension du fonctionnement des agences de l’eau. Cet ensemble, n’ayons pas peur de le dire, sème le doute sur la capacité des élus, des collectivités ou des chambres consulaires à gérer la politique de l’eau et remet en question leur légitimité.

Pour mieux gérer la ressource, une simplification du labyrinthe s’impose. En ce qui concerne la gestion quantitative de l’eau, nous devons bien évidemment prioriser l’accès à l’eau potable, puis notre souveraineté alimentaire. Pour ce qui est de l’accès à l’eau potable, le constat est sans appel : le volume d’eau perdue à cause des réseaux d’eau potable fuyards s’élève à 1 milliard de mètres cubes par an. Il est urgent de mobiliser les moyens nécessaires pour assumer nos responsabilités dans ce domaine. L’ampleur de cette perte, que l’on peut rapprocher de l’indispensable indépendance alimentaire, relativise le

Vous le voyez, madame la ministre, les enjeux relatifs à l’eau sont nombreux. C’est pourquoi, comme je l’avais recommandé dans un rapport en 2015, nous avons besoin d’une

La France doit relever le défi d’une gestion de l’eau durable et tournée vers l’avenir. Travaillons ensemble pour faire de cette politique de l’eau une priorité, sans idéologie, sans dogmatisme, mais avec pragmatisme. Bravo ! Mes